Madame la Première ministre, mesdames, messieurs les ministres, mes chers collègues, j'ai le plaisir de saluer, dans la tribune d'honneur,

La délégation est accompagnée par notre collègue Nadia Sollogoub, présidente du groupe d'amitié France-Ukraine, dont je veux saluer l'extraordinaire engagement en cette période.

Elles jouent un rôle crucial dans l'accueil des populations déplacées et l'organisation de la résistance. Elles témoignent de l'unité de la nation ukrainienne.

Ces crimes imprescriptibles devront être jugés, comme j'ai eu l'occasion de le souligner lors de mon déplacement à Kiev, afin de témoigner- le mot prend tout son sens -de la solidarité du Sénat à l'égard des autorités et du peuple ukrainiens. Les collectivités territoriales françaises se sont mobilisées, dès la première heure, pour venir en aide à l'Ukraine agressée : elles ont, dans un puissant élan de solidarité, accueilli des réfugiés participé à des convois humanitaires. Cet élan de solidarité fait honneur à notre pays. Le développement des relations entre les collectivités françaises et ukrainiennes, qu'il s'agisse de partenariats ou de jumelages, permettra d'ancrer dans la durée les liens de solidarité entre nos deux pays,

pour la liberté et la souveraineté retrouvée de leur pays. L'ordre

madame la Première ministre, mesdames, messieurs les ministres, mes chers collègues,

La 38 campagne des Restos du Coeur s'est ouverte hier, avec d'ores et déjà un constat : ceux-ci accueilleront 12 % de personnes en plus par rapport à l'année dernière. Au travers de mon intervention, je souhaite aborder plus généralement la question de la précarité alimentaire, qui touche, d'après le Secours populaire français, plus de 7 millions de nos concitoyens. Face à cette crise, le secteur associatif essaie de pallier les manquements de l'État. Malgré la solidarité qui s'organise, le contexte économique fragilise les associations

Cette même augmentation des prix de l'alimentation conduit à une baisse des dons des particuliers. C'est donc toute la chaîne de solidarité qui se trouve en difficulté.

Je veux d'ailleurs rendre hommage aux élus locaux présents dans nos tribunes et au congrès des maires, qui savent prendre leurs responsabilités, écouter, accompagner toutes tous pour leur apporter la réponse dont ils ont besoin. Cependant, les budgets des communes sont de plus en plus contraints par les politiques d'austérité conduites par le Gouvernement. Face à ce constat, il n'y a qu'une question : quand allez-vous prendre la mesure de l'urgence sociale qui touche notre pays ?

au-delà des 140 milliards d'euros qui ont déjà été mobilisés dans le cadre de différents dispositifs- mise en place du bouclier énergie, remises à la pompe ... -, le Gouvernement continue à accompagner les acteurs de l'aide alimentaire. La première loi de finances rectificative a prévu un effort exceptionnel de plus de 50 millions d'euros en faveur de l'aide alimentaire et des associations fragilisées par la hausse des prix des denrées. Elle a prévu, par ailleurs, le déblocage d'une enveloppe exceptionnelle de 10 millions d'euros de crédits d'aide alimentaire

novembre dernier, la création d'un fonds spécifique pour l'aide alimentaire durable, doté de 60 millions d'euros lors de son amorçage, en 2023, afin de renforcer, au-delà de la quantité, la qualité de l'aide alimentaire.

vous vous satisfaites de ce constat, tandis que, parallèlement, les patrons du CAC 40 ont doublé leurs revenus ! Je ferai toujours partie de celles et de ceux qui combattent les inégalités pour donner sens et coeur à la devise de notre République, « Liberté, Égalité, Fraternité

La présence des services publics dans nos territoires, particulièrement dans les territoires ruraux, est au coeur de bien des échanges dans les allées du 104 Congrès des maires de France. À mon tour, je veux saluer ici celles et ceux qui s'emploient sans relâche à améliorer le quotidien de nos concitoyens.

Autant de programmes que l'Agence nationale de la cohésion des territoires (ANCT) anime et pilote depuis leur lancement. Je puis ici témoigner de la qualité du travail mené par tous les acteurs. L'exemple de la ville de Douai, toujours dans le Nord, est à cet égard révélateur de la méthode partenariale mise en oeuvre, qui se concrétise par de premiers résultats salués par toutes et tous et par l'envie d'aller plus loin dans la redynamisation du territoire. La création de 200 brigades de gendarmerie, partout sur le territoire, grâce à la loi d'orientation et de programmation du ministère de l'intérieur (Lopmi), participe de ce grand mouvement, et l'attente des maires est grande, comme nous avons pu le vérifier le 7 novembre dernier, encore une fois dans le Nord, à Solesmes, sur l'invitation du ministre de l'intérieur. Là aussi, ce travail a pour vocation d'être mené dans un souci de partenariat, de mutualisation et donc d'efficacité, au service de nos concitoyens. Monsieur le ministre, il n'est pas de bonne série qui ne connaisse pas de suite, et les programmes gérés par l'ANCT n'échappent fort heureusement pas à cette règle. C'est notamment le cas du programme Action coeur de ville, dont la prochaine saison est attendue avec grande impatience après le succès du premier. Sobriété foncière, rénovation thermique et mobilité verte sont autant de défis qu'ont à relever nos collectivités, et la transition écologique est sans conteste- l'issue de la COP27 en témoigne -la priorité des priorités.

Monsieur le ministre, au lendemain de la tenue des 5 Rencontres nationales Coeur de ville, pouvez-vous nous détailler les priorités et moyens mis en oeuvre pour conforter, encore et toujours plus, l'impact de ces dispositifs dans les villes moyennes et, plus globalement, à l'échelle du territoire ? La parole

Je vous remercie de mettre en avant ces programmes si chers à la Première ministre et au Président de la République que sont Action coeur de ville, Petites Villes de demain et les maisons France Services. J'avais d'ailleurs eu l'occasion d'inaugurer l'une des premières maisons de ce type avec le Président de la République, à Amiens, il y a quelques années. Les programmes

Monsieur le président, madame la Première ministre, mes chers collègues, sur le plan financier, le climat entre l'exécutif et les collectivités territoriales est mauvais. Chaque début de quinquennat voit revenir les mêmes méthodes. Après la taxe d'habitation, vous vous attaquez aujourd'hui à la En 2022 comme en 2017, votre formule reste la même : aucune négociation réelle avec les associations d'élus. La main de l'État recentralisateur s'abat sans que les principaux concernés aient leur mot à dire.

Il n'est pas acceptable de fragiliser les collectivités, plus particulièrement les communes, qui ont souvent pallié les carences de l'État lors des crises précédentes. Il n'est pas acceptable non plus d'opposer artificiellement la dépense publique, qui pour vous ne serait qu'une charge, à la richesse créée par les entreprises. Les collectivités territoriales créent également de la richesse par le dynamisme de leurs investissements. Elles créent des emplois de services pérennes, qualifiés et non délocalisables. Ces services publics de qualité sont un choix de société- le seul bien de ceux qui ne possèdent rien. La disparition programmée de la fiscalité locale, remplacée par des dotations aléatoires de l'État, est contraire au principe de libre administration des collectivités territoriales. Nos 500 000 élus locaux, serviteurs de la République, ont besoin de respect et de lisibilité. Aussi, dans sa sagesse et sa diversité, le Sénat s'est opposé à la suppression de la CVAE en début de semaine. Ma question est simple, madame la Première ministre : allez-vous revenir sur votre politique d'asphyxie fiscale de nos communes ? Allez-vous respecter le vote de la chambre des territoires ?

réalité aux polémiques. Depuis 2017, ne vous en déplaise, l'État a été au rendez-vous. Lors de la crise sanitaire, nous avons mobilisé 10 milliards d'euros pour soutenir l'action essentielle des collectivités. Face à l'explosion des prix de l'énergie, nous prenons des mesures fortes avec l'amortisseur électricité et avec le filet de sécurité pour les collectivités fragilisées. Elles ne concernent qu'une minorité ! Au total, ce sont 2,5 milliards d'euros qui doivent permettre aux collectivités de faire face à la flambée des prix de l'énergie. Je vous rappelle que près de 30 000 communes pourraient bénéficier, comme les ménages et les très petites entreprises, du bouclier tarifaire. Ces dispositifs ont été conçus avec les associations d'élus et les parlementaires ; ils pourront, le cas échéant, être adaptés pour répondre à toutes les situations. Monsieur le président Kanner, sans vouloir être désagréable, je suis obligée de vous rappeler que l'action menée depuis cinq ans contraste avec celle qui a été accomplie pendant le quinquennat de François Hollande.

De notre côté, pour la première fois depuis treize ans, nous augmentons la DGF. Pour défendre le pouvoir d'achat des ménages et renforcer la compétitivité des entreprises, nous avons décidé de supprimer la taxe d'habitation et nous souhaitons supprimer la CVAE. Ces baisses d'impôts au profit des ménages et des entreprises seront naturellement compensées par un autre impôt plus dynamique et plus stable : la TVA. Depuis qu'une partie de la TVA est versée aux collectivités, cette ressource donne largement satisfaction. Je n'ai jamais entendu un élu regretter la dynamique de cette taxe qui, vous le savez, permet d'offrir à des territoires fragiles la croissance par la consommation nationale. Au-delà des ressources et à la demande des associations d'élus, le Gouvernement a soutenu le maintien du mécanisme de revalorisation forfaitaire des bases fiscales, qui atteindra 7 % en 2023. Le gain est de 2,8 milliards d'euros pour les collectivités. Enfin, je le redis, nous ne laisserons aucune collectivité sans solution. Monsieur le président Kanner, je mesure pleinement les inquiétudes que la période peut susciter. Mais plutôt que de rajouter de l'inquiétude à l'inquiétude en tentant de faire oublier votre action passée, ... Ayez de la mémoire ! ... je vous invite à travailler avec le Gouvernement pour améliorer notre accompagnement

Madame la Première ministre, puisque vous n'avez pas été désagréable, je ne le serai pas non plus en rappelant les responsabilités qui étaient les vôtres lors du quinquennat que vous avez critiqué

Très honnêtement, votre réponse n'est pas satisfaisante. Votre choix est fait : vous sacrifiez les collectivités territoriales La parole est à Mme Véronique Guillotin, pour le groupe du Rassemblement Démocratique et Social Européen. d'État chargée de la citoyenneté, en cette semaine de congrès des maires, et alors que nous accueillons au Sénat un grand nombre d'élus, ma question porte sur l'insécurité à laquelle ils sont trop souvent confrontés. Puisque l'actualité nous a tragiquement rappelé que cette insécurité touchait tous les représentants de l'autorité publique, j'aimerais avoir une pensée pour l'inspecteur des finances publiques qui a été lâchement assassiné lundi dans l'exercice de ses fonctions. Pour une part croissante de la population, le service public s'apparente de plus en plus à un bien de consommation courante, ce qui entraîne incivilités et agressions envers les représentants de l'État et des collectivités territoriales. Les chiffres le confirment : plus de 1 800 procédures judiciaires ont été engagées depuis janvier dernier pour des atteintes aux élus. Un chiffre en hausse constante, mais toujours en deçà de la réalité puisque la plupart des victimes ne portent pas plainte. les agressions à l'encontre de ceux qui se dévouent pour leur collectivité, souvent au détriment de leur vie personnelle et professionnelle. Comme le dit si justement le président Larcher, « à portée de baffe », particulièrement dans les petites communes qui manquent de moyens, les maires et les adjoints sont obligés d'intervenir eux-mêmes dans des situations parfois déjà tendues. Ces insultes, menaces et agressions physiques mettent l'élu et sa famille dans une situation d'insécurité inacceptable, et contribuent au nombre croissant de démissions. Le groupe RDSE, par la voix d'Éric Gold et Nathalie Delattre, a déposé deux propositions de loi sur ce sujet depuis 2019. La deuxième, adoptée récemment à l'unanimité au Sénat, prévoit la possibilité pour les assemblées et associations d'élus de se constituer partie civile au pénal pour soutenir un élu, ou l'un de ses proches, victime d'agression, de dégradation de bien ou de divulgation d'informations privées.

Même si cette COP a conduit au lancement d'un fonds spécifique pour répondre aux pertes et dommages des pays les plus vulnérables, elle n'a pas permis d'avancer vers un scénario crédible de stabilisation du réchauffement climatique sous les 2 degrés. En effet, alors que la COP de Glasgow avait appelé à une réévaluation des engagements des États, très peu sont venus en Égypte avec de nouvelles propositions. En remontant très légèrement son propre objectif, qui est de-57 % en 2030 au lieu de-55 %, l'Union européenne a néanmoins rappelé son rôle moteur dans cette négociation. Cet objectif européen nous engage et nous oblige à une réduction massive de nos émissions. Cette réduction passe nécessairement par la mobilisation des territoires, en particulier au travers des plans climat-air-énergie territoriaux, les PCAET. a d'ailleurs voté hier, à la quasi-unanimité, la mise en place d'une dotation climat systématique sur la base de 10 euros par habitant, pour permettre au bloc communal d'accélérer la transition écologique.

êtes-vous prête à entendre le message unanime que le Sénat a exprimé dans son vote d'hier, pour transformer une partie du fonds vert en une dotation climat annuelle systématique, qui donnera enfin aux territoires de véritables moyens de fonctionnement pour assurer leur transition et qui permettra à la France d'atteindre ses objectifs climatiques ?

il maintient l'objectif de limiter le réchauffement climatique à 1,5 degré. Réaffirmer cet objectif était nécessaire dans un contexte mondial de crise énergétique où la tentation aura été grande de renoncer. L'Union européenne, avec l'objectif de-57 % des émissions en 2030, que vous avez rappelé, montre la voie au niveau mondial. Nous, Français et Européens,

Vous m'interrogez sur les moyens que nous mettons au service de nos objectifs climatiques, en particulier sur le fonds vert. Ce fonds est un outil inédit en matière de financement de la transition écologique : il est entièrement dédié aux collectivités territoriales et traduit notre conviction

Les priorités ont été arrêtées sur la base des échanges que nous avons eus avec les collectivités et les services de l'État dans les territoires. Il s'agit, par exemple, de la rénovation des bâtiments publics, du recyclage des friches, du soutien au tri et à la valorisation des biodéchets, remplacement de l'éclairage public, de la renaturation des villes, ou de l'accompagnement à la mise en place de zones à faibles émissions (ZFE). Les remontées du terrain sont prometteuses : les collectivités se montrent intéressées par cet outil et nos échanges lors du salon des maires le confirment. Les préfets et les services déconcentrés sont prêts aussi à se saisir de cet outil dès le 1 janvier prochain. Monsieur le sénateur, le fonds vert est une dotation annuelle pour financer l'action des collectivités en faveur de la transition écologique.

à la veille du, période au cours de laquelle les échanges commerciaux s'intensifient, je souhaite vous alerter sur les dangers d'un nouveau vecteur de la contrefaçon, les influenceurs, sur la nécessité de lutter contre leurs pratiques illicites sur les réseaux sociaux. Si le volume de la contrefaçon est difficile à évaluer, s'agissant d'une activité clandestine par nature, la Cour des comptes estime raisonnable, pour 2019, de parler de 10 milliards d'euros de pertes fiscales pour l'État et de plus de 40 000 emplois détruits chaque année. Le phénomène de la contrefaçon, qui a connu un essor considérable au cours de cette décennie, menace potentiellement toutes les entreprises, fragilisant leurs efforts d'innovation et d'investissement et pillant leurs actifs immatériels. Il peut porter gravement atteinte à la sécurité des consommateurs, lorsqu'il concerne des médicaments, des pièces détachées automobiles ou des jouets. Il a également un impact néfaste sur l'environnement. Depuis peu, les réseaux sociaux, médias incontournables du marketing numérique, offrent un nouveau cadre à la contrefaçon. La simplicité d'utilisation de ces supports donne l'occasion aux internautes mal intentionnés de promouvoir et de commercialiser des produits de contrefaçon en toute discrétion. En effet, l'utilisation de ces médias, grâce notamment à la fonctionnalité des au caractère éphémère, permet aux influenceurs-contrefacteurs de proposer à la vente des produits de contrefaçon dont ils assurent la promotion, à l'insu des titulaires de droits. de droits. La France ne dispose toujours pas d'une stratégie nationale de lutte contre la contrefaçon, malgré les recommandations de la Cour des comptes. Face à la croissance exponentielle d'une nouvelle forme de contrefaçon sur les réseaux sociaux, pouvez-vous nous indiquer les mesures que vous envisagez de prendre afin de lutter activement contre le phénomène des influenceurs-contrefacteurs

Monsieur le ministre, elle s'appelait Vanesa, elle avait 14 ans. Ce vendredi 18 novembre, elle rentre du collège pour rejoindre le domicile de ses parents

violée, étranglée par un individu connu de la justice pour des faits antérieurs, commis lorsqu'il avait 15 ans. Il avait alors été condamné à quinze jours d'emprisonnement, assortis d'un sursis avec mise à l'épreuve de deux ans. Il n'était astreint à aucun contrôle judiciaire, à aucun contrôle par un service d'insertion et de probation.

interpellé. Le Lot-et-Garonne est en deuil, un deuil d'autant plus insupportable que c'est la troisième fillette qui est enlevée sur le chemin de l'école. Elle s'appelait Vanesa, elle avait 14 ans. Monsieur le ministre, c'est davantage la vice-présidente de La Mouette, association de protection de l'enfance, qui vous interpelle, et plus qu'une question, c'est un appel au secours.

pour que les associations de protection de l'enfance puissent mener à bien leur principale mission, la prévention, afin de sauver notre bien le plus précieux, la vie de nos enfants

Avec pudeur et émotion, au nom de notre assemblée, je tiens tout d'abord à exprimer notre solidarité aux parents de Vanesa. Je les ai rencontrés. Ce sont des gens admirables, qui sont venus dans notre pays pour travailler. Ils y ont malheureusement trouvé ce qu'il y a de pire pour des parents ... Face à l'horreur, ce sont toujours les mêmes questions qui reviennent : que s'est-il passé ? Cela aurait-il pu être évité ? À qui la faute ? Ces questions, je me les pose je vous les pose. Mais en passant en revue les circonstances du drame, il est bien difficile d'y répondre. S'agit-il d'un problème d'immigration ou de radicalisation ? Pas du tout, l'auteur présumé des faits n'a rien d'un étranger fiché S. S'agit-il d'une faute de la gendarmerie ? Absolument pas. Les gendarmes ont été très réactifs et ont immédiatement pris la situation au sérieux. S'agit-il d'une insuffisance des moyens municipaux de sécurité ? Encore moins. J'en sais quelque chose, c'est moi qui ai fait installer les caméras à Tonneins. Bien sûr, des voix ne manqueront pas de s'élever pour réclamer toujours plus de caméras, toujours plus de surveillance. Mais jusqu'où pousser la surenchère ? Ne risque-t-on pas de basculer dans une société dont personne ne veut ? Alors, il reste une dernière piste, que ma collègue a évoquée. l'assassin présumé avait déjà commis une agression. N'y a-t-il pas eu un défaut de suivi psychologique, médical et judiciaire, même si les faits remontent à seize ans ? Monsieur le ministre, qu'en pensez-vous et qu'allez-vous faire pour que de tels faits ne se renouvellent pas ? La parole

Je connais les profondeurs noires des esprits humains et les ravages que peuvent provoquer certains troubles mentaux. Je ne crois pas, mais l'enquête le dira, que l'état de cette personne était de nature à justifier un suivi psychologique ou psychiatrique. En tout cas, ce n'est pas ce qui avait été décidé lorsqu'il avait 15 ans. Cependant, vous l'avez dit vous-même, c'était il y a seize ans.

Honnêtement, je n'en suis pas sûr, mais sans les éléments complets de l'enquête il m'est difficile de vous répondre sur ce point. Néanmoins, sachez que la détermination des services de justice et de police, ainsi que du Gouvernement et de la représentation nationale, est totale, non pas pour comprendre ce que nos cerveaux humains ne peuvent pas comprendre, mais pour faire en sorte qu'un tel drame n'arrive plus jamais.

Le Sénat, dans le cadre de l'examen du projet de loi de finances, jouera son rôle pour essayer d'élargir le champ des communes éligibles au filet de sécurité. Notre inquiétude ne s'arrête pas là, madame la Première ministre. Nous sommes aussi inquiets de vos propos lorsque vous appelez, finalement,

Ma question, madame la Première ministre, est très claire : croyez-vous encore en la France communale ? Si tel est le cas, nous attendons, comme les maires, des preuves d'amour.

Il est au rendez-vous pour les aider et pour maintenir leurs capacités d'investissement. Il agit en concertation avec les associations d'élus pour coconstruire les solutions au plus proche du terrain. Vous pouvez aussi faire confiance aux anciens maires que nous sommes, Caroline Cayeux, Christophe Béchu et moi-même, pour être particulièrement attentifs à ces questions. Vous avez bien changé ! Nous sommes nous aussi des élus locaux attachés à nos territoires.

l'État soutiendra aussi les collectivités locales, en particulier les plus fragiles, face à la hausse du prix des énergies, grâce aux différents boucliers tarifaires que nous avons mis en place. Plus d'un milliard d'euros seront destinés

Nous avons en partage, madame la Première ministre, cette volonté de prêter plus d'attention aux actes qu'aux mots. C'est bien de cela qu'il s'agit et nous attendons

La parole est à Mme Victoire Jasmin, pour le groupe Socialiste, Écologiste et Républicain.

pour le bien vivre ensemble, trop souvent mis à mal dans ces territoires éloignés, en raison d'une défiance originelle à l'égard de l'État et de l'autorité. Or les collectivités territoriales d'outre-mer, qui pâtissent déjà d'un sous-financement chronique, d'une masse salariale très importante et d'un coût de la vie supérieur de 30 %, doivent, elles aussi, faire face à l'inflation sur les matières premières et sur l'énergie. C'est dans ce contexte de grande tension que le Gouvernement a consenti à des efforts supplémentaires en faveur du budget des outre-mer. Bien qu'insuffisants, ils sont néanmoins appréciables, pour peu qu'ils soient intégralement utilisés aux outre-mer fonde ainsi l'une des mises en garde du récent rapport de la Cour des comptes, qui demande que les engagements de l'État soient mieux suivis, avec un appui en ingénierie locale, en vue d'une meilleure utilisation des crédits alloués aux collectivités d'outre-mer.

d'excuser l'absence de mon collègue Jean-François Carenco, qui est actuellement avec le Président de la République au salon des maires, auprès d'élus ultramarins. Permettez-moi ensuite de témoigner de la solidarité du Gouvernement à l'égard du conseil régional de Guadeloupe,

les contrats de redressement en outre-mer (Corom), dits aussi contrats Patient-Cazeneuve- saluons le sénateur Georges Patient pour ce travail -, qui ont été lancés en 2021. Le dispositif, comme vous le savez, vise à accompagner les communes ultramarines faisant face à des difficultés financières. Neuf communes contractantes se sont engagées à optimiser leur gestion et à fiabiliser leurs comptes : il s'agit de Sada à Mayotte, Saint-Benoît à La Réunion, Cayenne et Iracoubo en Guyane, Pointe-à-Pitre, Saint-François et Basse-Terre en Guadeloupe, ainsi que Fort-de-France et Saint-Pierre à la Martinique. Il s'agit d'un partenariat gagnant-gagnant, la collectivité s'engageant sur une trajectoire financière de redressement et d'amélioration de gestion, l'État apportant des subventions de fonctionnement si les engagements sont tenus. Je veux vous rassurer sur un point : l'autonomie du maire est pleinement respectée, l'État ne faisant que l'accompagner dans la mise en oeuvre de ces contrats. La vague de contrats en cours est dotée de 30 millions d'euros répartis sur la Nous pouvons, par ailleurs, répondre à votre volonté d'élargir ces contrats à plus de communes, puisque l'Assemblée nationale a voté 30 millions d'euros supplémentaires pour les Corom en 2023. Cela nous permettra d'amplifier ce dispositif d'accompagnement des collectivités, qui, nous le croyons, fait largement consensus et je vous remercie de l'avoir rappelé dans votre question. Vous le voyez, madame la sénatrice, le Gouvernement agit et continuera de travailler, sous l'autorité de la Première ministre, en lien avec les maires ultramarins, pour accompagner leur volonté d'assurer une gestion saine de leurs finances, meilleur moyen de leur donner des marges de manoeuvre supplémentaires dans l'exercice de leur mission auprès de nos concitoyens d'outre-mer.

une réunion dite « convention des partenaires », consacrée à l'avenir de la Nouvelle-Calédonie. En cette circonstance, vous avez rappelé avec raison que, à l'issue du processus référendaire, l'avenir appartenait aux Calédoniens et qu'il leur revenait d'élaborer un projet d'avenir consensuel. Pour y parvenir, vous avez proposé la mise en place de groupes de travail, que le ministre de l'intérieur et des outre-mer doit installer lors de sa visite à Nouméa dans les jours prochains. Cette initiative est utile, puisqu'elle s'inscrit dans le choix que la Nouvelle-Calédonie a fait de rester française. Mais est-elle suffisante ? Les référendums de 2018, 2020 et 2021 ont ravivé les tensions et les divisions, réduisant en miettes cette « exception calédonienne » symbolisée par la fameuse poignée de main de main entre Jacques Lafleur et Jean-Marie Tjibaou en 1988. De partenaires, madame la Première ministre, nous sommes redevenus des adversaires. J'en veux pour preuve l'absence des mouvements indépendantistes à cette convention dite « des partenaires ». Et pourtant, pour élaborer ce projet d'avenir consensuel que vous appelez vous-même de vos voeux, nous n'avons pas d'autre choix que de renouer ces liens de confiance, car notre avenir ne se construira pas l'un sans l'autre ni l'un contre l'autre. Madame la Première ministre, concrètement, quelles initiatives le ministre de l'intérieur envisage-t-il de prendre lors de son séjour à Nouméa pour que les trois partenaires qu'étaient l'État, les indépendantistes et nous-mêmes, se retrouvent en confiance ?

de la convention des partenaires, qui s'est réunie le 28 octobre dernier, à la demande de la Première ministre. Vous étiez d'ailleurs présent. Comme vous le savez, le lancement de la convention des partenaires a marqué le début des discussions sur l'avenir institutionnel de la Nouvelle-Calédonie au terme du processus politique prévu dans l'accord de Nouméa. Le processus de définition d'un projet pour la Nouvelle-Calédonie, qui consacre sa place dans la République française et respecte ses singularités, est désormais engagé. Si les échanges du 28 octobre ont été denses et fructueux, ils sont restés incomplets, et vous en avez été le témoin, monsieur le sénateur, en raison notamment de l'absence d'une partie des forces politiques. Or, pour que le processus que nous avons engagé aboutisse, toutes les forces politiques calédoniennes doivent y contribuer. Le ministre de l'intérieur et des outre-mer se rendra donc en Nouvelle-Calédonie, accompagné du ministre délégué chargé des outre-mer, pour prendre le temps du dialogue et de l'écoute, afin que tous les partenaires politiques participent aux discussions dans un esprit de responsabilité et de consensus. Dans cette démarche, monsieur le sénateur, le Gouvernement sait qu'il pourra compter sur votre engagement personnel et sur votre capacité à nouer le dialogue avec les responsables indépendantistes, mais les discussions ouvertes par la convention des partenaires ont également vocation à traiter de sujets stratégiques pour l'avenir des Calédoniens. Au-delà des sujets institutionnels, qui feront l'objet de discussions, plusieurs groupes de travail seront organisés sur les sujets suivants égalité des chances et cohésion sociale, développement économique, emploi, grands investissements, nickel, souveraineté énergétique et transition écologique, souveraineté alimentaire, foncier, valeurs, identité commune et réconciliation, intégration et rayonnement régional. Dans ce contexte, le déplacement du ministre lui permettra également de rencontrer la société civile, la jeunesse, les acteurs économiques ou associatifs de Nouvelle-Calédonie, afin de comprendre les enjeux et les attentes, et de faire en sorte qu'ils puissent contribuer à la définition d'un projet qui intéresse d'abord l'ensemble des Calédoniens.

la situation des droits et libertés des femmes dans le monde est extrêmement préoccupante. En Afghanistan, les talibans nient les femmes ; en Ukraine, des femmes sont violées et subissent des violences sexuelles de l'envahisseur russe en République démocratique du Congo, en Syrie, en Éthiopie, en République centrafricaine, au Soudan, au Yémen, en Birmanie, le viol est utilisé comme arme de guerre. Les minorités yézidie, ouïghoure ou kurde ne sont pas plus épargnées.

Dans le cas de l'Iran, nous pouvons et nous devons agir, mais nous ne le faisons pas ou pas assez. L'Iran préside actuellement la commission onusienne de la condition de la femme ... Quel cynisme ! Notre collègue Marie-Arlette Carlotti a déjà soulevé ce paradoxe, le 9 novembre dernier. Le Gouvernement s'est dit impuissant : avons-nous été impuissants quand la Russie a attaqué l'Ukraine ? Non, nous ne nous sommes pas résignés Contre l'Iran, les sanctions n'empêchent pas la violence envers les manifestants. « Femme, Vie, Liberté » : madame la ministre, le slogan des femmes iraniennes impose à la France de s'élever contre la barbarie des mollahs et cela passe par la dénonciation de la présidence de cette commission onusienne de la condition de la femme par l'Iran. Qu'attendez-vous ? Quand cesserez-vous de mettre un voile sur la condition des femmes en Iran ?

Vie, Liberté » : face aux aspirations légitimes des Iraniennes et des Iraniens, le régime a choisi la voie de la répression, ce que nous avons condamné et continuons de condamner de la façon la plus claire. on recense de nouvelles victimes- plus de 300 déjà ! -, des jeunes femmes, comme Mahsa Amini, 22 ans, des enfants, comme Kian Pirfalak, 9 ans. Et cela dure depuis dix semaines À ces morts, il faut ajouter les arrestations, les détentions, la censure et les pressions contre les artistes, les avocats, les journalistes ou les simples citoyens. La France soutient les aspirations des Iraniennes et des Iraniens à plus de liberté. Le Président de la République a rencontré, le 11 novembre dernier, plusieurs Iraniennes exilées,

Notre action se décline dans toutes les enceintes internationales, qu'il s'agisse de l'Union européenne, qui a pris des sanctions à plusieurs reprises contre les responsables de la répression, de l'ONU, dont le Conseil des droits de l'homme, demain, jeudi, examinera la situation en Iran et créera un mécanisme d'établissement des faits pour que la vérité puisse être dite. Nous serons vigilants aussi, madame la sénatrice, pour que l'Iran ne puisse pas détourner la commission de la condition de la femme des Nations unies de son objet. Enfin, nous continuerons de demander nous continuerons de demander à l'Iran de cesser la répression, de respecter le droit de manifester pacifiquement et, bien sûr, de libérer immédiatement nos compatriotes retenus en otage. Et la question

à Mme la ministre déléguée chargée des collectivités territoriales, qui est absente. L'article 72 de la Constitution garantit la libre administration des collectivités territoriales, donc des communes, cellules de base de la démocratie. vues « d'en haut », les communes ne seraient qu'un échelon administratif, alors que, dans les faits, et on l'a constaté pendant la crise du covid-19, les communes et leurs élus se sont tenus au plus proche de nos concitoyens, en première ligne. à quoi assiste-t-on depuis plusieurs années ? À une véritable mise sous tutelle des maires qui, malgré de prétendues lois de décentralisation, ne disposent plus d'aucune autonomie fiscale. L'État a progressivement supprimé les impôts locaux, dont les communes fixaient librement le taux, pour les remplacer par des dotations et des impôts nationaux partagés. Et que dire des fameux contrats de Cahors et du mal nommé pacte de confiance, que le Gouvernement veut imposer à toute force ? Comme le constate l'économiste Michel Cabannes, « la garantie constitutionnelle de l'autonomie financière n'est plus qu'une façade », et, comme le dit Philippe Laurent, vice-président de l'AMF : « Ce que veut l'État, au fond, c'est la suppression de la fiscalité locale. » Ce que les maires peuvent retenir, eux, c'est que ce jacobinisme et cette recentralisation de moins en moins déguisée dénotent le peu de considération que l'État a pour eux et le mépris dans lequel il les tient. Quand le Gouvernement se décidera-t-il à entreprendre une vraie réforme fiscale, qui redonnera dignité et confiance aux maires, premiers élus du peuple ?

sont quatre fois plus importants en France qu'en Allemagne, et deux fois plus que dans l'ensemble de la zone euro. Le ministre de l'industrie que je suis souhaite continuer à réindustrialiser la France, notamment dans cette période extrêmement compliquée de hausse des coûts de l'énergie. Oui, cela passe par une réduction des impôts de production locaux. Est-ce que, pour autant, nous affaiblissons les recettes des collectivités locales ? La réponse est non ! C'est faux ! Non, parce que, vous le savez, nous compensons cette baisse de la fiscalité par une part des recettes de la TVA, qui, permettez-moi de vous le rappeler, est plus dynamique que la CVAE. La TVA, depuis dix ans, c'est 3,5 % de hausse des recettes tous les ans, contre 2,5 % pour la CVAE. Mesdames, messieurs les sénateurs, les collectivités territoriales y gagneront. Est-ce que, pour autant, nous devons nous devons réduire les incitations des collectivités territoriales à la réindustrialisation ? La réponse est encore non ! Nous créons un fonds d'attractivité industrielle qui sera

Monsieur le ministre, le « pacte de confiance » désigne le nouveau dispositif de limitation des dépenses de fonctionnement des collectivités proposé par le Gouvernement. Derrière cette formule, on distingue très nettement l'esprit des contrats de Cahors, en pire ! Tant et si bien que, sur le terrain, il est renommé : « pacte de défiance La démarche du Gouvernement se vit dans les territoires, qu'ils soient de banlieue, urbains ou ruraux, comme une recentralisation diffuse du fonctionnement des collectivités territoriales, dont l'État grignote de plus en plus les prérogatives. La transformation des impôts locaux directs en compensations supprime la fiscalité dynamique des communes, entraîne une dépendance financière à l'égard de l'État et révèle la volonté sous-jacente de prendre la main sur les politiques locales. Cet état d'esprit jacobin remet en cause le principe constitutionnel de libre administration des collectivités. Alors que le Gouvernement se dit engagé dans un nouvel acte de décentralisation, les services de l'État, nationalement et localement, surinterprètent souvent les textes ou règlements, au détriment des exécutifs locaux. Auparavant, l'État accompagnait les maires pour réaliser leurs projets, mais nous sommes passés à la méthode de l'injonction ; désormais, nous en sommes à la contrainte. Les maires ne sont pas les simples exécutants des priorités de l'État. Monsieur le ministre, allez-vous favoriser l'accompagnement des collectivités, leur faire confiance et stopper cette mise à mal du principe de décentralisation voulu par la loi de 1982

on ne peut pas ! Le Gouvernement a fait le choix d'introduire le « pacte de confiance » dans le PLF pour 2023, sous la forme d'un rapport du Gouvernement au Parlement. Tous les acteurs publics, État comme collectivités territoriales, doivent participer à l'effort collectif pour rétablir les comptes de la Nation. Il y va de la crédibilité de notre pays à l'égard de nos partenaires européens. C'est le sens des trajectoires budgétaires inscrites en loi de programmation des finances publiques. Nous serons bien sûr attentifs aux débats qui se dérouleront ici, au Sénat, sur le sujet. Vous savez que le Gouvernement est à l'écoute des collectivités territoriales, donc de vous-mêmes, mesdames, messieurs

Elle sera territorialisée pour le bloc communal et forfaitisée pour les départements, comme je l'ai rappelé tout à l'heure. Enfin, il ne s'agit pas de réduire l'autonomie des collectivités. Nous passons d'un système de CVAE nationale,

du « qui décide paie, qui paie décide ». Si vous souhaitez réindustrialiser nos territoires et assurer la transition écologique de notre pays, il vous faut entendre les élus locaux, car vous ne pourrez pas faire sans eux. Ils demeurent incontournables, comme l'a démontré la gestion de la crise sanitaire. La parole est à Mme Catherine Belrhiti, pour le groupe Les Républicains. Monsieur le président, madame la Première ministre, chers collègues, la sécheresse historique de cet été nous rappelle combien la question de la gestion de la ressource en eau est essentielle pour notre pays. y répondre, le Sénat rendra cette semaine un rapport dans lequel nous définissons des priorités pour éviter de nous retrouver, demain, dans une situation encore plus difficile que celle d'aujourd'hui. Nous nous interrogeons toutefois sur la motivation du Gouvernement à agir concrètement et en phase avec les attentes des territoires. en matière de gouvernance, le Sénat s'est prononcé sur la nécessité de préserver la souplesse d'un transfert facultatif de la compétence en eau de la commune vers les intercommunalités, pour une raison très simple : l'eau répond à une logique de bassin versant et non de périmètre intercommunal.

et se voient ponctionner une part importante de leur budget, notamment par l'Office français de la biodiversité (OFB). De fait, comme cela a déjà été exprimé, nous redoutons que, contrairement au principe fondateur, l'eau ne paye plus l'eau, mais que l'eau paye l'État. Comme souvent, vos choix- ou plutôt votre absence de décisions -mettent à mal nos territoires. Ma question est donc simple, madame la Première ministre : entendrez-vous la voix des territoires, qui demandent plus de liberté dans la gouvernance de l'eau et plus de moyens pour agir ? M. le ministre délégué chargé de la ville et du logement.

Dans une période transitoire, qui doit permettre de laisser aux acteurs le temps de s'organiser, l'État gérera certains ouvrages jusqu'en 2024. Ce transfert représentera indéniablement des investissements importants pour les collectivités, ... Elles souffrent ! ... là encore, j'en sais quelque chose, puisque j'appartiens à un EPCI dont le bassin verse sur la Marne et que nous avons donc des obligations dans le cadre des jeux Olympiques de 2024- et nous les tiendrons ! Plusieurs outils financiers sont déployés pour les accompagner : le fonds de prévention des risques naturels majeurs (FPRNM) appuiera jusqu'en 2027 les études et les travaux sur les anciennes digues de l'État

loi 3DS, a ouvert une expérimentation destinée à mieux associer les établissements publics territoriaux de bassin à cette politique, par des financements dédiés. Elle permet également aux EPCI de se regrouper dans des structures dédiées afin d'atteindre la bonne échelle de gestion hydrographique. L'État accompagne donc les collectivités dans ce transfert et- cela a déjà été dit ici par mes collègues Christophe Béchu et Bérangère Couillard -sera très attentif à la gestion de l'eau et à la d'en disposer dans toutes les communes de France. Les moyens et les capacités financières ouverts sont donc importants, tout comme les leviers de gouvernance. La parole la réplique. Nous réaffirmons que la décision de transférer ou non la compétence de l'eau vers un syndicat ou une intercommunalité doit rester celle de la commune. Par ailleurs, sans préservation des moyens de financement des agences de l'eau, il est inenvisageable de relever les défis de demain en matière de gestion de la ressource ; le pire est à redouter. Encore un domaine dans lequel les collectivités territoriales se sentent sacrifiées.

Le Gouvernement souhaite un dialogue apaisé avec les élus, mais un nouveau signal complètement inverse leur a été envoyé dans le projet de loi de finances en cours d'examen. En effet, lors des débats à l'Assemblée nationale, le Gouvernement a déposé, discrètement, un amendement tendant à revenir sur les modalités de la participation de l'État et de France compétences au financement de l'apprentissage dans la fonction publique territoriale.

Cet accord, conclu en octobre 2021 et unanimement salué par les associations d'élus, a fait l'objet d'une signature officielle au mois de janvier dernier et a été intégré dans le code général de la fonction publique.

Madame la ministre, nous avons vraiment du mal à nous y retrouver ... Les budgets sont déjà compliqués à boucler- nous l'avons déjà évoqué. Si les engagements de l'État bougent au gré du vent et au gré des ministres, comment voulez-vous que les collectivités s'engagent avec assurance dans un tel processus de recrutement d'apprentis ?

par la loi Élan, à la TFPB au titre de locaux professionnels. Or la seule activité de ce type d'habitat est de loger des personnes souvent âgées et seules, souhaitant privilégier un cadre convivial. Les services à la personne proposés dans les parties communes de ces lieux ne sont pas exercés par les bailleurs, lesquels ne tirent pas de rémunération dans ce cadre. Dès lors, pour quelle raison leurs loyers devraient-ils relever de la taxe foncière au titre d'une activité professionnelle ? C'est tout un modèle économique vertueux qui est ainsi menacé : l'habitat inclusif constitue une solution résidentielle

madame la ministre, le nouvel abattement sur délibération de taxe foncière sur les propriétés bâties que vous proposez ne manquerait pas d'être revendiqué par d'autres contribuables tout aussi dignes d'intérêt, ce qui risquerait d'affecter directement les ressources des collectivités concernées. L'efficacité L'efficacité du dispositif semble incertaine, dans la mesure où l'abattement serait attribué au bénéfice du seul propriétaire, sans que soit prévue, en contrepartie, une déduction du loyer mis à la charge du résident. Il n'est pas certain que l'allégement de TFPB

Or elle constitue un atout majeur dans la lutte contre ce changement climatique, car elle est à la fois un puits de carbone et un réservoir de biodiversité. En France, trois millions de propriétaires détiennent une ou plusieurs parcelles forestières d'une superficie inférieure ou égale à 4 hectares. Certains propriétaires ne savent même pas qu'ils le sont ; d'autres n'envisagent pas la gestion de leur parcelle du fait d'une trop petite superficie. En réalité, l'extrême fragmentation des parcelles de terrain empêche la bonne gestion de la forêt, notamment la mise en place d'actions de protection de la biodiversité et de valorisation économique économique et écologique. Cet amendement vise ainsi à encourager les propriétaires forestiers détenant de petites parcelles à confier la gestion de leur propriété à un groupement forestier en instaurant, d'une part, un montant minimal de taxe foncière pour les parcelles de terrain en nature de bois et forêt d'une superficie inférieure ou égale à 4 hectares et, d'autre part, en exonérant de taxe foncière sur les propriétés non bâties les propriétaires de ces parcelles qui rejoindraient un groupement forestier. La parole

madame la ministre,

conduirait à mettre en place deux systèmes de calcul d'imposition pour une seule et même taxe. Elle présenterait ainsi un risque de rupture d'égalité devant la loi et les charges publiques. L'objet de ces amendements se trouve par ailleurs en opposition avec des dispositifs qui ont été institués en matière de taxe foncière sur les propriétés non bâties en faveur des espaces naturels, agricoles et forestiers. En cohérence avec les objectifs de protection de la biodiversité, les terrains ensemencés, plantés ou replantés en bois, les terrains boisés présentant un état de futaie irrégulière en équilibre de régénération sont en effet exonérés. En réalité, une telle mesure conduirait à plus de complexité dans la gestion de la fiscalité directe locale, sans pour autant que son efficacité soit assurée. En effet, l'application d'un montant minimal de 13 euros de taxation ne paraît pas susceptible de susciter des ventes ou des regroupements de parcelles. être complète, la mise en place de bonnes pratiques de gestion forestière relève plus de dispositifs non fiscaux, à l'instar d'outils de planification tels que le programme national de la forêt et du bois ou les schémas régionaux de gestion sylvicole. Pour toutes ces raisons, le Gouvernement demande le retrait de ces amendements madame la ministre,

Mme Raymonde Poncet Monge. Cet amendement vise à conditionner l'exonération de la taxe foncière octroyée aux terrains ensemencés, plantés ou replantés en bois à des conditions permettant d'assurer une sylviculture plus proche des cycles naturels. D'une part, il tend à mettre fin aux coupes rases de complaisance conduisant au remplacement d'un peuplement existant par une nouvelle plantation, alors que des itinéraires techniques d'amélioration à moindre impact sont possibles. D'autre part, il tend à favoriser la diversification des peuplements et donc la résilience des forêts au changement climatique, en cohérence avec la feuille de route du ministère de l'agriculture pour l'adaptation des forêts au changement climatique.

À cette fin, la libre évolution peut être prévue par une obligation réelle environnementale, en particulier si la totalité de la parcelle est concernée. Le propriétaire peut aussi bénéficier de cette exonération s'il dispose de garanties de gestion durable au sens du code forestier, c'est-à-dire s'il existe un document de gestion forestière ou que le propriétaire adhère au code de bonnes pratiques sylvicoles. Ne sont donc pas concernées les propriétés laissées à l'abandon. Cette exonération présente un double intérêt : elle favorise la libre évolution tout en incitant les propriétaires à l'ancrer dans un cadre de gestion contrôlé. Si les surfaces en libre évolution ont attiré l'attention, raison de leur intérêt pour la biodiversité. En effet, les arbres âgés, le bois mort sous toutes ses formes et les écosystèmes caractéristiques des forêts en libre évolution sont les supports de vie d'un quart de la biodiversité terrestre. Ils abritent notamment certains prédateurs participant à la lutte contre les parasites. Ces espaces sont, par ailleurs, un laboratoire d'observation précieux pour l'adaptation au changement climatique, au sein duquel s'expriment des mécanismes de régulation naturelle.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

être attentifs à préserver des ressources pour les collectivités territoriales. Je ne suis pas persuadé qu'une exonération de taxe

et à permettre aux communes qui le souhaitent de mettre en place un régime d'accompagnement vers cet état en profitant d'une exonération de la part communale de cette taxe pendant cette période transitoire. En effet, la futaie irrégulière ou foresterie à couvert continu présente de nombreux intérêts en matière de lutte contre le changement climatique, de préservation de la biodiversité, de production de bois de qualité et d'acceptation sociale. En s'appuyant naturellement sur un mélange d'essences, d'âges et de structures au sein d'une même forêt, cette forme de sylviculture, peu développée en France, répond aux enjeux de nombreuses politiques publiques et doit donc être encouragée. La conversion à une sylviculture à couvert continu implique, pour de nombreux propriétaires, de faire appel à une expertise extérieure et d'engager des travaux dont le coût est supérieur aux recettes qu'ils peuvent espérer à court terme. À ce titre, et puisque ces travaux concourent à atteindre des objectifs de politiques publiques relatives au climat et à la biodiversité, un accompagnement fiscal

exercent une mission de santé et d'intérêt public auprès des personnes fragiles sans logement. La nouvelle mise en oeuvre de la taxe d'habitation, au regard du volume global du budget des établissements concernés, représente en moyenne 2 % à 4 % d'augmentation,

d'où notre inquiétude. En réalité, ce sont surtout les 20 % des ménages les plus aisés qui verront leur pouvoir d'achat augmenter de près de 1 200 euros, alors que de nombreuses autres familles continuent de se battre pour boucler les fins de mois. La taxe d'habitation n'était déjà pas payée par les Français les moins aisés : les 16 % de foyers les plus modestes en étaient exonérés. Cette réforme ne leur profitera donc pas, contrairement aux 20 % de foyers les plus riches, qui gagneront en moyenne 1 158 euros et capteront 44,6 % des 17,6 milliards de coûts pour le budget de l'État de cette réforme. Quel

Le calcul de cette compensation intègre un coefficient correcteur pondéré par deux facteurs, visant une répartition juste et équitable au sein du département en fonction du produit fiscal perçu par la commune avant 2020. Toutefois, dans les départements ruraux, les montants de la taxe foncière dépassent en volume ceux de la suppression de la taxe d'habitation. L'excédent collecté par les contribuables des communes dudit département se trouve ainsi réaffecté à d'autres collectivités, essentiellement urbaines et souvent plus aisées. plus aisées. Ce sont donc des ressources provenant des communes rurales, moins favorisées, qui viennent compenser des communes souvent plus urbaines, où le pouvoir d'achat est plus élevé et où la contribution à la solidarité fiscale peut donc se faire sous une forme différente. Ce changement de calcul permet ainsi de majorer le coefficient correcteur. Cette majoration vise à supprimer les effets de bord du mécanisme de compensation, où les communes rurales participent de manière disproportionnée à l'effort fiscal. Il s'agit donc de rétablir une péréquation

pour les contribuables, comme pour les parlementaires, tous deux introduits sur mon initiative. L'article 42 dispose en effet que soit précisé sur les avis d'imposition le montant de la retenue sur le produit de la TFPB ou du versement complémentaire résultant de l'application du coefficient correcteur, afin que le contribuable puisse connaître la part de cet impôt qui n'est pas mobilisable pour le financement des services publics de sa commune, au titre du dispositif national de compensation de la suppression de la taxe L'article 43 avance quant à lui d'un an, soit au 1 mars de l'année prochaine, la remise du rapport du Gouvernement au Parlement sur les conséquences sur le schéma de financement des communes concernant la suppression de la taxe d'habitation sur les résidences principales. Ces deux observations conduisent la commission à émettre un avis défavorable

Depuis la mise en place de la réforme de la taxe d'habitation et du coefficient correcteur, certaines communes ont constaté une erreur dans le calcul du coefficient, le plus souvent liée à une erreur de déclaration d'un contribuable en 2020, exemple pour conséquence une hausse importante du foncier bâti déclaré. Ainsi, le coefficient correcteur notifié est inférieur à ce qu'il aurait dû être, ce qui entraîne notamment des pertes de recettes parfois très substantielles pour le budget de petites communes. Dans ces cas de figure, la DGFiP, qui a constaté les difficultés, explique qu'elle ne peut recalculer le coefficient, car aucune disposition légale ne permet de procéder à ce retraitement.

L'objet de cet amendement est de permettre que, en cas d'erreur, le coefficient correcteur pour neutraliser l'impact financier du remplacement de la taxe d'habitation par la taxe sur le foncier bâti

? Chacun le sait, le coefficient correcteur a pour objectif de faire correspondre l'ancienne part départementale de la taxe foncière avec la ressource de taxe d'habitation « perdue » par la commune dans le cadre de la réforme de la suppression de la taxe d'habitation. Cela permet de calculer la ressource dynamique de compensation pour la commune. L'une des lignes importantes de la réforme, c'était que ce coefficient était calculé

en permanence pour 36 000 communes, on imagine l'impact en matière de gestion pour les services de la direction générale des finances publiques. L'amendement vise à donner la possibilité de corriger le coefficient pour des communes où il y aurait eu une erreur. De ce point de vue, l'esprit de l'amendement est satisfait, puisque, aujourd'hui, en cas d'erreur importante, une commune peut tout à fait faire un recours gracieux auprès de la DGFiP

On va regarder cela de près, monsieur le sénateur ! S'il faut rappeler la doctrine à l'ensemble des services de la DGFiP pour leur dire que, lorsqu'il y a un recours parce qu'il y a une erreur, il faut revoir

la loi de finances pour 2020, revirement de situation : plutôt qu'un dégrèvement assumé par l'État, le Gouvernement choisit la part de taxe foncière sur les propriétés bâties des départements. Les taux de la taxe d'habitation étant figés à ceux de de préciser que les communes perdantes ont été assez nombreuses. Il y a eu des gagnantes et des perdantes, des communes sous-compensées et d'autres surcompensées, car les périmètres de ces deux impôts n'étaient pas équivalents. C'est à ce moment-là que le Gouvernement a eu l'idée de mettre en place un coefficient correcteur, le fameux « coco », qui n'a aucune relation avec l'étiquette de notre groupe. Ce dispositif illisible a vocation à s'appliquer aux communes surcompensées qui ont perçu plus de taxe foncière que ce à quoi elles auraient pu prétendre dans le cadre de la taxe d'habitation.

Reichardt. Le code général des impôts prévoit une exonération de la taxe foncière sur les propriétés non bâties (TFPNB) pour les terrains situés dans un site Natura 2000 faisant l'objet d'un engagement de gestion.

L'introduction d'un coefficient de minoration à partir de 2009 a ainsi progressivement fait supporter aux communes rurales l'entier coût des mesures socles de mise en oeuvre de la politique Natura 2000, à savoir les contrats Natura 2000 et les chartes correspondantes.

Je rappelle qu'une compensation intégrale à 100 % de l'exonération de la taxe foncière est possible pour les communes et les EPCI dont le budget de fonctionnement est touché à plus de 10 %. %. À ma connaissance toutefois, il n'existe pas de communes ou d'EPCI dont le montant de l'exonération de la taxe foncière sur les propriétés non bâties représente au moins 10 % du budget de fonctionnement.

de sens que s'il s'agit d'une mesure générale. Il est compliqué de le faire dans des cas particuliers, même si l'on entend bien l'objet de vos amendements et les territoires que vous visez, monsieur le sénateur. La compensation de certaines exonérations de fiscalité locale, parmi les plus anciennes, fait l'objet de minorations dans le cadre de variables d'ajustement qui sont l'un des instruments permettant d'assurer la maîtrise des concours financiers de l'État aux collectivités. C'est le cas de la compensation de l'exonération de taxe sur la TFPNB pour les sites Natura 2000, qui est prévue depuis 2006. Il faut rappeler que, dans un contexte de crise, le Gouvernement a cherché à limiter le plus possible ces minorations en retraitant les hausses des concours financiers intervenues en 2020 et 2021 et liées à la crise. Ces variables atteignent depuis cette année un niveau très faible ; en 2021 et en 2022, leur montant atteint 50 millions d'euros contre 182 millions d'euros en moyenne entre 2013 et 2020. Il n'est pas prévu d'exclure la compensation de l'exonération de TFPNB sur les sites Natura 2000 de l'assiette des variables. Néanmoins, je rappelle que les sites Natura 2000 bénéficient de la dotation biodiversité, laquelle participe au verdissement des concours de l'État aux collectivités locales. Elle a vocation à accompagner les communes dont une part du territoire est classée dans une zone visant à la protection de la biodiversité et qui sont, à ce titre, soumises à un certain nombre de charges. Instituée en 2019 sous le nom de dotation Natura 2000, pour un montant de 5 millions d'euros, elle a été renommée une première fois en 2020 en tant que dotation biodiversité, ce qui accompagnait, d'une part, le doublement de ce montant, passé ainsi à 10 millions d'euros-

une attente très forte des communes concernées, qui, à l'heure actuelle, sont obligées de faire face seules aux contraintes créées par Natura 2000 dans les différents sites, ce qui est tout à fait injustifiable. C'est la raison pour laquelle je ne peux pas retirer ces amendements,

Malgré un réexamen de l'amendement n° I-1696 rectifié, on voit mal juridiquement comment on peut moduler le mécanisme de variable d'ajustement qui est un mécanisme général.

la tarification incitative sur une partie seulement de leur territoire et supprime le délai d'harmonisation des modes de financement du service public de gestion des déchets. Ce changement législatif éviterait les difficultés techniques rencontrées par les collectivités locales, qui ont des territoires très différents : les collectivités pourraient ainsi déployer la tarification incitative sur la partie de leur territoire qui se situe en milieu périurbain et rural et ne pas être obligées de le faire en milieu urbain où le déploiement peut paraître plus complexe. Cet amendement vise à donner de la souplesse aux élus locaux, qui connaissent les réalités de leur territoire, pour adapter la tarification des déchets en fonction des freins et des opportunités.

des ordures ménagères (Teom) et perdent ainsi le caractère incitatif de la fiscalité des déchets. Or ces territoires sont souvent des pionniers de la tarification Il serait particulièrement préjudiciable que des années d'efforts de la part d'élus locaux volontaires soient remises en cause par une simple limite juridique. La Cour des comptes a par

soit la taxe d'enlèvement des ordures ménagères, soit la redevance d'enlèvement des ordures ménagères sur une partie de son territoire. Dans la mesure où la dernière modification

les résultats de cette première étape de modification avant de modifier à nouveau le dispositif existant, et ce pour une raison assez simple : il est

l'effort consenti sur un territoire. À juste raison, monsieur Kern, vous avez évoqué le fait que le dispositif de redevance est plus souvent pratiqué dans les territoires ruraux peu denses,

Aujourd'hui, ce plafonnement est égal à 100 % de la valeur locative moyenne. Cet amendement vise à le ramener à 50 % de la valeur locative moyenne.

n° I-929 rectifié. Depuis le début de nos travaux, nous avons été nombreux à faire part de notre ambition pour les territoires, singulièrement pour les communes, en leur apportant davantage de souplesse pour qu'ils puissent mieux répondre aux attentes de leurs habitants et au souci de leur gestion. L'objet de cet amendement s'inscrit dans cette manière de voir il ne coûte rien à l'État et il n'impose rien aux collectivités. La taxe d'enlèvement des ordures ménagères s'appuie sur les bases fiscales du foncier bâti, dont on sait qu'elles sont totalement désuètes- nous en avons longuement parlé ce matin.

mais il ne me semble pas nécessaire de contraindre plus étroitement les communes ou les intercommunalités dans la définition

à offrir aux villes la possibilité d'instaurer une Teom incitative à une échelle collective. En clair, la tarification serait basée sur des flux de déchets mesurés collectivement par secteur, les secteurs pouvant être des communes, des quartiers, des îlots ou des immeubles. Il s'agit de donner une liberté supplémentaire aux collectivités territoriales.

pour que les maires, en particulier dans les secteurs urbains, puissent conjuguer les vertus environnementales de la taxe incitative et l'efficacité des mesures de secteur.

Après l'adoption de la loi NOTRe et à la suite des fusions de territoires menées en 2017, de nombreuses communautés nouvelles présentent aujourd'hui, sur leur périmètre périmètre intercommunal, des modes de financement différents pour leur service des déchets. Cette variété de régimes fiscaux sur un même territoire a été rendue possible par le législateur qui, tout en visant un objectif d'harmonisation, a permis le maintien d'une coexistence de modes de financement antérieurement choisis par les communes ou EPCI fusionnés, et ce pendant un délai de sept ans. Ce délai dérogatoire avait pour objet de permettre aux EPCI de faire des choix de politique fiscale harmonisés et vertueux, en prenant le temps de la réflexion et en permettant des transitions fiscales acceptables pour les usagers du service public des déchets. Cette expérience a permis aux EPCI concernés de constater les bienfaits du maintien de modes de financement diversifiés sur leur territoire. Le présent amendement a donc

Plus de 4 milliards de personnes utilisent des décharges illégales ou non réglementées, qui accueillent 40 % des déchets. Et 5 % des émissions de gaz à effet de serre dans le monde sont dues à la décomposition et au traitement des déchets. La gestion des déchets dans les pays en développement constitue donc un enjeu environnemental majeur et présente une importante marge de progression, pourtant peu mise

Nous avons une part importante de responsabilité dans tous les déchets que nous produisons et que nous ne traitons pas en France. Prévoir ce 1 %, c'est une petite action que nous pouvons mener,

pour la protection du pouvoir d'achat, cet amendement vise à assurer un plafonnement de l'augmentation de la taxe foncière à 4 % et non à 7 % comme envisagé par le Gouvernement.

C'est un comble que l'État décide de supprimer une taxe revenant aux collectivités et oblige ces mêmes collectivités à en augmenter une autre. Cela s'appelle dépenser l'argent des autres, monsieur le ministre

Cet amendement vise à décaler la hausse du plafond de la taxe foncière de 2023 à 2024, afin de préserver le pouvoir d'achat des ménages encore concernés par la taxe d'habitation, qui représentent 20 %

vise à moduler le taux de la taxe de publicité foncière ou du droit d'enregistrement, aujourd'hui fixé à 3,80 %. Ce dernier peut être modifié par les conseils généraux sans que ces modifications puissent avoir pour effet de le réduire à moins de 1,20 % ou de le relever au-delà de 4,50 Nous proposons un dispositif de droits de mutation plus égalitaire avec la mise en place d'un barème progressif qui taxerait moins les acquisitions inférieures à 200 000 euros, et davantage les transactions plus importantes, tout en conservant le même niveau de recettes

Les départements ont perdu leur dernier levier de fiscalité propre, la taxe foncière, en conséquence de la suppression de la taxe d'habitation et de la mise en place d'un mécanisme de fiscalité partagée.

Il s'avère encore plus pertinent aujourd'hui à l'aune de la crise énergétique, du retour de l'inflation, de la hausse des prix des carburants et de la nécessité de réduire l'autosolisme.

augmenter le plafond du versement mobilité que les collectivités territoriales ont la faculté d'instituer pour financer leurs transports publics.

la compétence d'autorité organisatrice de la mobilité de disposer d'un surcroît de ressources pour soutenir leurs services publics de transport.

Je comprends donc la volonté des auteurs de ces amendements. Néanmoins, je le dis franchement, je suis réservé sur la solution qu'ils préconisent, qui conduirait à accroître la pression fiscale sur nos entreprises,

atteinte. Je demanderai donc l'avis du Gouvernement sur l'ensemble de ces amendements. Je voudrais m'assurer que l'exécutif a pris toute la mesure de la gravité de la situation et connaître les solutions qu'il entend

collègues, la situation de l'établissement est critique. Si l'on ne fait rien, Île-de-France Mobilités pourrait n'avoir d'autre choix que de réduire son service,

Rappelons-nous qu'en loi de finances rectificative pour 2020, dans le contexte de début de crise sanitaire, des avances remboursables de l'État avaient été accordées à Île-de-France Mobilités.

les solutions à mettre en oeuvre ne peuvent être prises sans l'organisation d'une vaste concertation. C'est d'autant plus vrai que les opérateurs franciliens devront bientôt faire face au défi de l'organisation des jeux Olympiques de Paris 2024. C'est la raison pour laquelle je proposerai, en seconde partie de PLF, un amendement prévoyant d'organiser dès le premier trimestre 2023 une conférence une conférence du financement des transports publics en Île-de-France. Celle-ci serait chargée de mettre sur la table des solutions permettant de soutenir efficacement l'établissement face à la crise,

C'est d'autant plus vrai que cet impôt pèse déjà très largement sur les entreprises franciliennes- nous sommes un certain nombre dans cette enceinte à le savoir. Celles-ci contribuent à hauteur de 45 % au financement des transports publics, sans compter l'obligation pour les employeurs de financer 50 % des abonnements de transports en commun de leurs salariés.

Il y a selon moi des questions à se poser sur le modèle. Le versement mobilité représente 40 % des ressources d'IDFM. Il n'est pas tenable, de notre point de vue, d'augmenter sans cesse les impôts de production pour aboutir,, à un modèle

1 % d'économies sur le fonctionnement, c'est 100 millions d'euros d'économies ! Je redis la disponibilité du Gouvernement dans son ensemble, et plus particulièrement de la Première ministre et de mes collègues Christophe Béchu et Clément Beaune, pour continuer de travailler sur ce sujet avec les élus de la région Île-de-France. En ce qui concerne les autres amendements, vous aurez compris pourquoi nous sommes défavorables à une augmentation du versement mobilité.

mais nous ne pouvons pas nous contenter de ce constat. Si on ne peut faire autrement, c'est parce que le besoin d'investissement existe aussi dans les transports en commun et dans les transports collectifs. On est en train d'imposer des zones à faibles émissions dans les grandes agglomérations. Il faut donc développer des alternatives aux véhicules

est l'implication des entreprises dans les transports publics. Nous sommes l'un des seuls pays où les entreprises sont directement associées au financement des transports publics. Que ce soit en Allemagne, en Espagne, en Italie, aux États-Unis ou au Canada,

d'euros de subventions, 750 millions d'euros d'avances remboursables et derrière cela, un plan mobilité de plus de 3,5 milliards d'euros.

la validation de cet amendement, c'est la santé financière de la métropole qui serait remise en question. Nous ouvririons une crise institutionnelle majeure au sein de cet ensemble, qui représente, je vous le rappelle, quatre fois le Grand Paris et six fois le Grand Lyon. Quel

fléchés sur le budget transports de la métropole. Nous vous proposons un déplafonnement progressif et régulé. Des simulations ont été faites pour lever uniquement 80 millions d'euros, ce qui

le nombre d'usagers des transports est le même qu'avant la pandémie, on n'a retrouvé nulle part le niveau de trafic suffisant : il manque des rames, il manque des métros, il manque des RER.

du matériel, pas assez d'argent pour embaucher- on manque de chauffeurs et de conducteurs -, pas assez d'argent pour investir dans la formation. Il faut donc trouver des recettes supplémentaires. On peut tourner autour du pot, mais c'est absolument indispensable.

sur les usagers alors que la situation dans les transports est aujourd'hui totalement dégradée. de la vie quotidienne de millions de personnes, qui vivent une situation extrêmement dégradée. Tous les jours, des missions, des bus, des métros, des RER

J'ai répondu à l'invitation de la présidente de la région Île-de-France, qui n'est pas exactement une amie politique, parce qu'elle a attiré l'attention sur le grave danger, pour Île-de-France Mobilités d'une impasse financière de 950 millions d'euros. Je m'adresse à toutes les travées

je soutiens la proposition qu'a formulée Mme Pécresse d'une hausse du versement mobilité modulée selon la richesse. Quand on paie son siège social ou son siège d'entreprise à La Défense ou dans le coeur de Paris, excusez-moi, mais ce n'est pas le montant du versement mobilité qui va nuire à l'équilibre budgétaire de l'entreprise ! Nous avons une nécessité ardente de répondre aux besoins des usagers et je serais étonné, chers collègues, que vous ne soyez pas solidaires avec votre présidente de région.

pour permettre le voiturage des athlètes et des journalistes. Voilà un surcoût énorme, qui est à la charge d'Île-de-France Mobilités et qui n'est pas financé par l'État.

le ministre ? Quand il n'y aura plus un seul conducteur de bus volontaire, nous aurons fait beaucoup d'économies de fonctionnement, mais nous n'aurons pas résolu les problèmes des transports publics.

explication de vote. Monsieur le ministre, ce que je regrette dans tout cela, c'est qu'on a l'impression que l'État est ailleurs.

Jean-Paul Huchon avait alors fait venir Manuel Valls, Premier ministre, qui avait pris un certain nombre d'engagements sur le financement par l'État des transports publics en Île-de-France. Ces engagements n'ont pas été respectés.

D'autres ont dit que l'État fuyait ses responsabilités. Pourtant, le rapport de la Cour des comptes dit qu'il y a eu, ces trois dernières années, « une intervention massive et inconditionnelle de l'État » pour Île-de-France Mobilités.

ou « virtuel » pour bénéficier de l'exonération. Plus fondamentalement, je pense que le versement mobilité doit être considéré non comme une redevance, mais bien comme un impôt, assis sur la masse salariale, permettant de financer les transports publics, dont- je le répète -il me semble peu opportun de fragiliser les recettes dans le contexte actuel. La commission demande donc le retrait

une évaluation des principales caractéristiques des bénéficiaires de l'exonération de forfait social pour les versements abondant les contributions des salariés sur les plans d'épargne entreprise

contradiction avec l'objectif affiché de développement des opérations d'actionnariat salarié pour le plus grand nombre. D'autre part, cela pourrait conduire à attribuer un avantage fiscal

Si les clients ont eu le choix d'accepter ou non le transfert de leurs produits financiers vers la nouvelle banque, avec laquelle l'ancienne avait passé un accord, il n'en a pas été de même pour leur contrat d'assurance vie. En effet, comme vous le savez, il est actuellement impossible pour un client de transférer son contrat d'assurance vie vers l'entreprise d'assurance de son choix, sauf à fermer son contrat, donc à perdre les avantages fiscaux liés à sa date d'ouverture.

parfois avec des prélèvements automatiques, se retrouve dans une situation étrange. Il peut ouvrir des comptes auprès de n'importe quelle institution financière, mais il ne peut rien faire pour son contrat d'assurance vie. On l'oblige même à aller vers la banque ou l'assurance choisie par l'ancien

Plus de 420 000 contrats ont ainsi été transférés en 2021. Le dispositif prévu par la loi Pacte, qui est utilisé en pratique, nous paraît suffisant pour répondre aux besoins des épargnants.

telle transférabilité représenterait un choc de nature à dégrader les ratios de solvabilité des assureurs vie français. Ensuite, renforcer la transférabilité des contrats d'assurance vie diminuerait la contribution de l'assurance vie au financement des entreprises françaises, ainsi que le rendement de l'épargne.

En effet, malgré le rachat de HSBC Bank par My Money Group, les contrats restent gérés par HSBC Assurances. De même, la fin des activités d'ING en France n'a pas entraîné un changement d'assureur

à l'imposition forfaitaire sur les entreprises de réseaux (Ifer). Le produit de cette imposition profite aux communes et aux conseils régionaux sur les territoires desquels ces centrales sont installées.

Cet amendement vise à porter ce montant à 24 euros par kilowatt de puissance installée. Pourquoi ? D'abord, les nuisances pour le voisinage, bien que limitées par rapport à d'autres types de centrales, n'en sont pas moins réelles. C'est d'ailleurs pour cette raison que le Gouvernement a soutenu la création du dispositif voilà quelques années. Surtout, il s'agit de tenir compte de la montée en puissance de la centrale et des résultats croissants de l'entreprise américaine qui l'exploite. Compte Compte tenu de la croissance de l'activité de cette entreprise, un tel taux ne serait nullement de nature à bousculer son équilibre financier et, plus précisément, sa marge bénéficiaire. En revanche, il représenterait une bouffée d'oxygène pour la petite commune de Bouillante. C'est pourquoi je vous invite, mes chers collègues, à adopter cet amendement. Quel

selon le principe : « 1 euro aux actionnaires, 1 euro aux salariés ». En effet, les mesures d'urgence pour le pouvoir d'achat doivent être accompagnées d'un élan plus ambitieux. Un meilleur partage de la valeur en entreprise entre l'ensemble des parties prenantes est ici un élément clé, à condition que les entreprises soient incitées à verser des enveloppes de participation suffisamment importantes.

campagne de mettre en place un dividende salarié, sur un fondement assez simple : quand l'entreprise verse des dividendes à ses actionnaires, elle doit aussi en verser à ses salariés. Il faut instaurer un mécanisme pour que, quand des dividendes sont versés aux actionnaires, les salariés soient immédiatement et directement intéressés. C'est un chantier que nous allons mener en 2023. Nous avons d'abord demandé aux partenaires sociaux d'en discuter et d'y travailler ensemble. Nous y travaillerons